La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du jeudi 24 octobre 2024 a été publié sur le site internet du Sénat. Il n’y a pas d’observation ?… Le procès verbal est adopté. J’ai le regret de vous faire part du décès de notre ancien collègue Guy Lèguevaques, qui fut sénateur de la Haute Garonne de 1996 à 1998,

Par lettre en date du 25 octobre, M. Patrick Kanner, président du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, a demandé que le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant la ratification de l’accord se rapportant à la convention des Nations unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, inscrit à l’ordre du jour du mardi 5 novembre soit examiné selon la procédure normale. Acte est donné de cette demande.

selon la procédure normale, soient examinés en troisième point de l’ordre du jour du 5 novembre et non en premier point, comme c’est actuellement prévu. Acte est donné de cette demande.

de cette demande. J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale est parvenue à l’adoption d’un texte commun. J’informe le Sénat qu’ont été publiées des candidatures pour siéger au sein de la commission spéciale sur le projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité.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 L’ordre du jour appelle le scrutin pour l’élection d’un juge suppléant à la Cour de justice de la République. Il va être procédé, dans les conditions prévues par l’article 86 du règlement, au scrutin secret pour l’élection d’un juge suppléant à la Cour de justice de la République. Ce scrutin se déroulera dans la salle des conférences ; la séance ne sera pas suspendue durant les opérations de vote. Je rappelle que la majorité absolue des suffrages exprimés est requise pour être élu. Une seule délégation de vote est admise par sénateur. Je remercie MM. Philippe Tabarot et Mickaël Vallet, secrétaires du Sénat, qui vont superviser ce scrutin. Je déclare ouvert le scrutin pour l’élection d’un juge suppléant à la Cour de justice de la République. Il sera clos dans une demi heure. Nous reprenons la discussion de la proposition de loi visant à assurer l’équilibre du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles. Dans la discussion générale, la parole est à Mme Christine Lavarde, auteur de la proposition de loi. Monsieur le

En effet, le changement climatique conduira à une augmentation certaine de la fréquence et de l’intensité des inondations, qui a déjà été constatée lors des dernières décennies.

La garantie de l’État n’a été appelée qu’une seule fois, en 2000, à la suite des tempêtes Lothar et Martin, et le taux de couverture contre les catastrophes naturelles en métropole est de 97 %.

nous constatons que ce régime est à bout de souffle. La provision pour égalisation de la Caisse centrale de réassurance va tomber à zéro à la fin de l’année et le risque que la garantie de l’État soit mobilisée est réel.

L’article 1 de la proposition de loi crée ainsi un mécanisme de revalorisation automatique annuelle du taux de la surprime pour tenir compte des effets du changement climatique. Celui ci doit permettre de lisser

a donc été adopté en commission pour assouplir le dispositif, en supprimant la condition du « même aléa naturel ». L’article 3 introduit une présomption de refus d’assurance pour le motif d’une exposition aux catastrophes naturelles dans les zones les plus à risque. Actuellement, la possibilité de saisine du bureau central de tarification est entravée par la difficulté pour les assurés de prouver que le refus d’assurance dommages aux biens est lié au risque CatNat. Dans le

envers cette profession et d’en renforcer l’attractivité, alors que les récents épisodes d’inondations ont souligné le manque d’experts qualifiés. L’article 5 instaure deux dispositifs distincts. D’une part, il rétablit la liberté d’utilisation des indemnités d’assurance en cas de sinistre provoqué par le phénomène de retrait gonflement des argiles. D’autre part, il impose à l’assureur, lorsque celui ci établit que le phénomène de RGA constitue la cause déterminante d’un sinistre, de notifier cette information au maire de la commune

Si nous partageons l’objectif de l’article 5, un retour à une liberté totale d’affectation des indemnités versées en RGA ne nous paraît pas opportun, notamment au regard du risque de fraude. Les assurés peuvent en effet effectuer des travaux superficiels et vendre le bien. Il nous a donc semblé souhaitable de maintenir le principe d’affectation en prévoyant deux exceptions claires : lorsque le coût des réparations excède la valeur du bien et lorsque le bâtiment est devenu inhabitable. C’est le sens de l’amendement que nous avons adopté en commission. en commission. L’article 6 créait un dispositif de modulation de la franchise en cas d’adoption de mesures de prévention par les assurés. Si nous partagions l’objectif de cet article, à savoir le renforcement de la culture du risque chez les particuliers,

de l’expérimentation « Mieux reconstruire après inondation ». Cette identification des travaux nécessaires intervient en complément de l’article 7, qui crée un dispositif incitatif de soutien à l’acquisition de prêts pour la prévention des risques,

8 conditionne l’octroi de MaPrimeRénov’ à la réalisation de travaux de prévention des risques pour les logements les plus exposés. Pour paraphraser Jean Marc Jancovici, qui s’est exprimé sur

d’un enjeu de cohérence avec la politique d’adaptation au changement climatique. Enfin, l’article 9 étendait le champ du fonds pour la prévention des risques naturels majeurs à des dispositifs expérimentaux retrait gonflement des argiles et du recul du trait de côte. Le risque RGA concerne près de la moitié des logements individuels et il n’existe aucun soutien public de grande ampleur à sa prévention. De plus, ce risque est assuré dans le cadre du régime CatNat. concerne le recul du trait de côte, il s’agit d’une question majeure, mais le fait qu’il ne soit pas couvert par le régime CatNat peut poser des difficultés techniques à son intégration dans le champ du fonds Barnier.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, entre 2020 et 2025, la sinistralité liée aux catastrophes naturelles devrait augmenter de 47 %.

Si nous voulons continuer à honorer ce principe constitutionnel, dans un contexte d’intensification de la sinistralité et de montée en charge du risque retrait gonflement des argiles, nous devons impérativement adapter notre régime d’indemnisation des catastrophes naturelles. C’est

à répondre aux besoins futurs. La commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, conformément à son champ d’expertise, s’est concentrée sur le volet prévention des risques, qui est central pour garantir la pérennité du régime.

L’article 11, inspiré d’une recommandation du rapport d’information relatif aux inondations survenues en 2023 et au début de l’année 2024, s’inscrit dans cette continuité. Le cadre scolaire me semble en effet propice au développement d’une conscience de la réalité des risques et à l’apprentissage des pratiques à adopter pour mieux les prévenir.

l’obligation de réaliser une étude géotechnique dite G1, au stade de la cession du terrain ou de la construction du logement. Les études G1 sont toutefois très limitées selon les données que nous ont fournies les administrations, elles ne sont parfois qu’un plagiat des données nationales. Dans certains cas, elles sont même réalisées par des professionnels peu scrupuleux, dépourvus de toute qualification technique. Oh là… Au stade de la construction, le particulier peut soit recourir à une étude G2,

Il est bien plus efficient de généraliser ces études géotechniques que de financer la réparation des bâtiments endommagés. Je forme le vœu que, pour les ménages les plus modestes, le surcoût puisse être pris en charge par la solidarité nationale, afin qu’aucun de nos concitoyens ne reste sur la touche. il me semble souhaitable que, lors de la vente d’un logement ou de la location d’un bien, l’acheteur ou le locataire ait connaissance de l’ensemble des risques. C’est le sens de l’article 12, qui fait figurer le risque de les informations devant être inscrites dans l’état des risques obligatoire, pour les logements situés dans une zone exposée au risque de sécheresse. En parallèle, l’article 8 vise à renforcer la prévention des risques tout au long de la vie des logements. L’Agence nationale de l’habitat (Anah) est chargée d’améliorer la qualité des logements. À ce titre, elle est notamment responsable du pilotage du programme de rénovation énergétique MaPrimeRénov’.

dans le Nord, dans le Sud Est, dans le Sud Ouest ou en région parisienne, le changement climatique entraîne et va continuer d’entraîner la multiplication de ces épisodes.

naturelles. Notre pays dispose d’un outil qui a fait preuve de son efficacité pour venir en aide aux personnes sinistrées : le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles. Ce régime, géré par la Caisse centrale de réassurance, a été créé en 1982. Reposant sur les principes de responsabilité, de solidarité et d’équité nationales entre citoyens et entreprises, il permet de couvrir les risques naturels de manière mutualisée.

qui améliore la prise en charge au profit des occupants, renforce la loi du 28 décembre 2021 relative à l’indemnisation des catastrophes naturelles, laquelle a déjà permis de mieux indemniser les assurés en cas de dommages liés aux catastrophes naturelles.

Le Gouvernement a également mené un travail de pédagogie, en détaillant par circulaire la procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle et les critères retenus pour chaque péril.

l’équilibre financier, il a annoncé une augmentation de la surprime « catastrophes naturelles » de 12 % à 20 % sur les contrats d’habitation, à partir du 1 janvier 2025. Cette hausse est nécessaire pour assurer la pérennité du régime et renforcer ses moyens d’action, mais elle n’est pas suffisante. En effet, dans un contexte marqué par des catastrophes naturelles plus fréquentes et plus intenses, il est primordial que les ressources du régime soient réévaluées régulièrement.

C’est pourquoi le précédent gouvernement a annoncé l’été dernier la création d’un observatoire de l’assurabilité des risques. Les travaux conduits par la Caisse centrale de réassurance permettront d’objectiver ce phénomène. En parallèle, le Gouvernement est en train de réaliser une cartographie des aléas naturels, pour éclairer l’observatoire et mieux informer le public à l’échelle des territoires.

Le fonds Barnier, qui constitue un pilier de notre politique de prévention, verra ses moyens passer de 225 millions à 300 millions d’euros par an à partir de 2025 – je tiens à

toujours le même objectif : mieux protéger les Français face aux catastrophes naturelles. Mes chers

Rééquilibrer le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles est une priorité pour nos territoires, comme pour la protection de nos concitoyens, particulièrement en cette période où les inondations affectent de nombreux départements de France.

D’autres dispositions méritent d’être saluées, comme l’augmentation du taux de surprime, qui introduit un mécanisme de réajustement en fonction des risques réels encourus. De même, le renforcement des garanties d’indépendance des experts est nécessaire pour rétablir un lien de confiance entre assureurs et assurés.

Aujourd’hui, la Gemapi est une compétence partagée de manière complexe et peu efficace. Les intercommunalités qui en sont chargées manquent de moyens face à l’ampleur des enjeux.

Nous devons agir ensemble, dans un cadre renforcé et simplifié, pour répondre efficacement à la menace grandissante des événements climatiques et mettre un terme au morcellement des compétences, qui ralentit gravement l’action publique en cas d’intempéries. Il est impératif d’alléger la contrainte législative pesant sur les travaux de curage. Le code de l’environnement limite le périmètre d’action des collectivités territoriales et empêche l’entretien de nos cours d’eau.

l’Histoire nous rappelle qu’il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Ah ! En simplifiant les processus administratifs, en renforçant les structures locales et en prenant pleinement en compte la problématique de la gestion des compétences, nous serons mieux armés pour protéger nos territoires.

renforcer le financement du régime, un mécanisme de revalorisation du taux de surprime, et mieux protéger les assurés lors de la procédure d’indemnisation, par l’encadrement de l’expertise et la lutte contre le phénomène de non assurance.

Certains territoires et certains biens ne seraient plus assurables à des tarifs abordables. Face à cette menace, les derniers gouvernements ont obtenu plusieurs avancées. L’ordonnance du 8 février 2023 a ainsi facilité la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour le phénomène de RGA. Afin de rééquilibrer le régime, le précédent gouvernement a également pris un arrêté augmentant la surprime CatNat. En conséquence, au 1 janvier 2025, le taux de la prime sur les contrats d’assurance « dommages aux biens » atteindra 20 %, contre 12 % actuellement.

l’article 9, qui étend le fonds Barnier au financement d’études et de dispositifs expérimentaux de prévention des dommages, la mention du recul du trait de côte a été supprimée.

Ces évolutions, nous ne les souhaitons pas à n’importe quel prix. Elles doivent s’inscrire dans la continuité de notre modèle, fondé sur la solidarité et la mutualisation, très protecteur, donc précieux.

Après les épisodes de crues et d’inondations qui ont gravement touché le département des Hautes Pyrénées au mois de juin 2013, les habitants de la ville de Lourdes ont ainsi pu obtenir 100 millions d’euros au titre des dégâts, quand les professionnels de l’hôtellerie et de la restauration bénéficiaient d’un soutien de 150 millions d’euros supplémentaires.

l’équilibre de notre système, son équité et son acceptation, on ne pourra se contenter de rehausser le taux de la surprime ou de renforcer le mécanisme de revalorisation automatique.

la déconnexion entre le produit de la taxe sur la surprime CatNat, finançant ce fonds, et le montant de celui ci. L’année dernière, le déséquilibre atteignait 73 millions d’euros.

une reconstruction à la fois plus rapide et plus résiliente des biens immobiliers des collectivités territoriales endommagés par une catastrophe naturelle. Cette logique

Mes chers collègues, vous l’avez compris, les élus du groupe RDSE sont particulièrement soucieux de soutenir nos territoires et nos concitoyens, de plus en plus malmenés par les aléas climatiques. Notre régime assurantiel doit répondre à ces cinq mots d’ordre : prévention, investissement, simplification, solidarité et adaptation.

Ces catastrophes naturelles, d’une violence extrême, ont bouleversé des vies, emporté des lieux de vie, des commerces et des souvenirs, laissé des familles, des entreprises et des territoires profondément meurtris. À tous ceux qui ont vu leurs biens et parfois le travail de toute une vie réduits à néant, j’adresse mes pensées les plus sincères et solidaires.

Que notre travail législatif aujourd’hui soit à la hauteur de la nécessité de mieux protéger nos concitoyens face à ces drames appelés à se multiplier. Les aléas naturels dommageables ont plus que quintuplé depuis les années 1970.

Face à ces risques, la solidarité nationale est une véritable nécessité. C’est tout l’intérêt de la proposition de loi que nous examinons aujourd’hui, puisque celle ci vise non seulement à améliorer l’assurance en matière de catastrophe, mais aussi à favoriser le développement de la prévention face aux risques naturels majeurs. Concernant la réforme de l’assurance des catastrophes naturelles, Centriste ne peut qu’encourager la mise en place d’un mécanisme de revalorisation automatique de la surprime. Nous partageons bien sûr le constat d’une crise de confiance entre assurés et compagnies d’assurances. Pour cette raison, nous soutenons aussi bien la suppression de l’application de la franchise multiple, en cas de succession d’aléas naturels sur une période courte, que l’instauration d’une présomption de refus d’assurance pour les biens situés dans les zones les plus à risque. groupe Union Centriste est également favorable à l’instauration de garanties d’indépendance vis à vis des experts d’assurance spécialisés dans les catastrophes naturelles et des experts d’assurés. De même, l’obligation de faire figurer dans le rapport d’expertise les préconisations des travaux de réduction de la vulnérabilité nous semble tout à fait pertinente. Enfin, nous jugeons particulièrement opportune la création de deux exceptions au principe d’affectation de l’indemnité d’assurance, à savoir dans le cas où le coût des réparations excède la valeur du bien et lorsque le bâtiment est devenu inhabitable.

Afin d’assurer l’équilibre du régime d’indemnisation, les efforts de prévention sont absolument nécessaires. Notre capacité à résister aux catastrophes naturelles à long terme repose largement sur la promotion d’une culture du risque qui sera généralisée. C’est pourquoi nous soutenons non seulement la mise en place d’un prêt à taux zéro pour financer les mesures de prévention, mais aussi l’extension du fonds Barnier au financement d’études et de dispositifs expérimentaux de prévention des dommages provoqués par les RGA.

finances a prévu une évaluation de l’impact de cette mesure sur la politique de rénovation énergétique. Il est nécessaire d’éviter les investissements publics inefficaces, sans nuire pour autant aux objectifs de rénovation énergétique des logements. Enfin et surtout, nous partageons la volonté des rapporteurs de promouvoir une véritable culture du risque. Je tiens d’ailleurs à saluer l’excellent travail de Pascal Martin, rapporteur pour avis de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. Ses amendements, repris par la commission des finances, enrichissent considérablement cette proposition de loi en ce qu’ils ont pour effet d’encourager le développement d’une conscience de la réalité des risques et des pratiques à adopter à tous les niveaux.

rééquilibrage des relations entre assurés et compagnies d’assurances, incitation à la prévention, réduction de la vulnérabilité du bâti et, surtout, promotion d’une culture du risque.

La fréquence des phénomènes climatiques étant inexorable, la transition est fondamentale pour les prévenir. L’adaptation, bien qu’essentielle, est un palliatif qui ne fera qu’amoindrir l’exposition des populations les plus vulnérables. Certes, elle limitera les dégâts, mais elle ne contribuera pas à maintenir la vie sur des territoires menacés. le Pas de Calais a connu trois épisodes d’inondations d’une violence inouïe, jamais vue de mémoire d’homme. Depuis le début du mois de novembre 2023, ce sont plus de 200 communes et plus de 450 000 habitants qui ont subi des épisodes de crues. Comme à chaque occasion, les habitants concernés se démènent pour sauver ce qui peut l’être et constatent, impuissants, les carences du système assurantiel : délais à rallonge, difficultés à justifier les pertes par des factures introuvables, démarches administratives lourdes et franchises onéreuses.

Il n’existe pas de civisme assurantiel. En effet, les assureurs profitent d’épisodes climatiques majeurs pour augmenter les tarifs des contrats d’assurance habitation, soit 115 euros supplémentaires dans une commune du Pas de Calais en proie aux inondations. Ajoutez à cela le quasi doublement de la surprime CatNat au 1 janvier prochain,

à l’universalité des surprimes sur tous les contrats de l’ensemble du territoire, cette proposition de loi est fondée sur la logique du chacun pour soi. La responsabilité individuelle supplante la responsabilité des assureurs. La collectivisation du risque climatique se heurte à la préservation de leur rentabilité. Aucune contribution nouvelle ne leur est demandée, rien sinon éviter la multiplication des franchises pour un même phénomène climatique. Les assurés doivent financer leur protection aux catastrophes naturelles : telle est la philosophie

Pourquoi la création d’un nouvel outil à l’article 7, sur le même modèle que l’éco PTZ, ne déboucherait elle pas sur un échec comparable ? Quant aux collectivités territoriales, elles sont absentes du texte : je le regrette. Elles ne semblent pas intéresser le Sénat, alors que 1 500 d’entre elles se trouvent en grande difficulté pour trouver

de sécurité nationale. On peut regretter que ce texte remette à demain les décisions que notre modèle assurantiel exige aujourd’hui pour se préparer à la multiplication et à l’intensification des phénomènes climatiques. La parole

madame la ministre, mes chers collègues, pour la seconde fois cette année, le Sénat examine un texte relatif au régime d’indemnisation des catastrophes naturelles. En préambule, je tiens à saluer la qualité des différents travaux menés au Sénat et notre engagement collectif à élaborer une réponse politique et efficiente à ces fléaux qui vont encore s’intensifier.

Le problème de financement du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles est réel. La Caisse centrale de réassurance (CCR) était déficitaire de 83 millions d’euros en 2023. Selon ses représentants, il existe de faibles chances qu’elle sollicite la garantie de l’État d’ici à la fin de l’année 2024. Cependant, elle estime que le coût de la sinistralité devrait augmenter de 40 % à l’horizon 2050. La mise en place d’un mécanisme de revalorisation s’impose donc.

touchés par des épisodes de sécheresse, donc de retrait gonflement des argiles, considérant qu’elle n’était pas financée et coûterait bien trop cher aux assureurs. Au travers de la

Mes chers collègues, voici le résultat du scrutin pour l’élection d’un juge suppléant à la Cour de justice de la République : Nombre de votants : 289 Nombre de suffrages exprimés : 242 Majorité absolue des suffrages exprimés : 122 Bulletins blancs : 44 Bulletins nuls : 3 M. Teva Rohfritsch a obtenu 242 voix. Ce candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, il est proclamé juge suppléant à la Cour de justice de la République.

Cozic. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, réchauffement climatique, sols argileux, acidification des océans, montée des eaux et destruction des littoraux, érosion des sols, pluies acides, fonte des glaciers, bouleversement du cycle de l’eau, inondations répétées… Je pourrais continuer longtemps à décliner la litanie

Il y a urgence à agir, tant nous observons une expansion géographique du risque de retrait gonflement des argiles, que le réchauffement climatique rend prégnant. Si nous nous projetons jusqu’en 2050, l’ensemble des coûts cumulés pourrait s’élever à près de 43 milliards d’euros, dont 17 milliards seraient directement attribuables aux seuls effets du changement climatique. Ce texte fixe plusieurs objectifs notables. Bien que perfectible, il a la volonté d’apporter une réponse politique au défi du réchauffement climatique et à la mécanique de hausse à venir des phénomènes de catastrophes naturelles, tout en garantissant aux citoyens une équité dans l’attribution des aides financières

1 ajuste automatiquement la surprime d’assurance pour mieux intégrer les impacts du changement climatique une réévaluation tous les cinq ans du régime CatNat. J’appelle votre attention sur le fait que la surprime CatNat est financée directement par les assurés au travers de leur contrat d’assurance. De fait, l’assureur applique un taux supplémentaire sur la prime d’assurance de base pour couvrir les risques de catastrophes naturelles. Cela signifie que chaque assuré contribue financièrement à ce système, même s’il ne vit pas dans une zone à risque.

lors de la répétition d’un même aléa naturel sur un territoire, et ce en généralisant une pratique déjà partiellement appliquée pour certains sinistres majeurs. Cette disposition est à mettre

La proposition de loi que nous étudions aujourd’hui vise à renforcer le régime CatNat. C’est un sujet d’une importance capitale pour la protection de nos concitoyens et de notre patrimoine national face aux risques climatiques qui, hélas ! se multiplient et s’intensifient. mois, le département du Nord a subi plusieurs épisodes d’inondations d’une grande ampleur, mettant des centaines de personnes et de familles en difficulté. Ce texte contient des dispositions que nous considérons comme positives et nécessaires, car elles vont dans le sens de la solidarité nationale, de la protection des biens et des personnes et du renforcement de la sécurité de nos territoires. Toutefois, nous exprimons de sérieuses réserves sur l’article 1, qui ne peut recevoir notre plein assentiment. Nous comprenons la logique d’équilibrer le texte en faveur des sociétés d’assurances, elles qui voient leurs obligations et charges augmenter par la création de nouveaux droits en faveur des assurés touchés par ces catastrophes.

du tout ! Les sociétés d’assurance, aujourd’hui largement bénéficiaires, peuvent et doivent participer davantage au financement d’un dispositif largement soutenu sinon par l’argent public, du moins par l’action publique. cette hausse automatique des primes est un obstacle. Si nous souhaitons garantir l’efficacité du régime d’indemnisation, cela ne doit pas se faire au détriment des assurés, qui risquent d’être accablés par des hausses constantes de leur cotisation. Nous défendrons donc un amendement visant à modifier une répartition juste du financement entre les assurés et les assureurs.

de loi améliore le financement du régime d’indemnisation en simplifiant les procédures, afin que les victimes obtiennent des remboursements plus rapides. C’est une demande que nous formulons depuis longtemps pour soutenir nos compatriotes dans les moments difficiles. Nous approuvons également l’article 2, qui limite les franchises appliquées aux sinistres successifs sur une période courte. Il s’agit là d’un geste juste et responsable pour ceux qui subissent plusieurs catastrophes rapprochées. ainsi protégés contre des frais supplémentaires qu’ils ne devraient pas avoir à supporter. L’article 4 va dans la même direction, en imposant une indépendance renforcée des sociétés d’expertise chargées d’évaluer les dégâts. Cette initiative garantit que les intérêts des assurés seront préservés et que les indemnisations seront calculées de manière juste et objective. Il est fondamental que ces experts soient libres de tout conflit d’intérêts avec les assureurs, si tant est que l’on veuille restaurer la confiance des Français dans le système d’indemnisation. Ainsi, mes chers collègues, nous soutiendrons les avancées de ce texte en matière de protection et de solidarité, mais nous appelons le Sénat à modifier l’article 1, afin que notre régime d’indemnisation demeure à la fois solidaire, juste et supportable pour l’ensemble des Français. La parole

la Seine et Marne, comme de nombreux départements français – de l’Ardèche au Nord, en passant par la Loire –, a subi de plein fouet, ces dernières années, et même ces derniers mois, l’augmentation à la fois en fréquence et en intensité des événements climatiques.

Ajoutons y les épisodes de sécheresse, notamment en 2023. Tout cela contribue, bien sûr, à fissurer les maisons, à endommager les fondations et à entraîner des réparations considérables,

Toutefois, la multiplication de ces événements pose nécessairement la question d’une réforme, ce que Mme la ministre n’a pas manqué de souligner. Quelles sont limites du dispositif actuel ? D’abord, la forte baisse des provisions d’égalisation, ensuite, les difficultés pour les communes d’obtenir la reconnaissance d’état de catastrophe naturelle,

Comment permettre à un système déjà fragilisé d’absorber, de prévenir les dommages actuels et ceux qui se produiront Cette proposition de loi de notre collègue Christine Lavarde – dont je salue l’excellent travail –, cosignée par de nombreux sénateurs, constitue une première étape

en renforçant notre résilience, en confortant le bâti, en adoptant des mesures de prévention et en finançant des dispositifs expérimentaux.

Il y a définitivement un avant et un après les 2 et 3 octobre 2020, tant cette tempête a durablement meurtri ces vallées.

Dans la suite de ces événements, j’ai été frappée de constater l’importance stratégique du fonds de prévention des risques naturels majeurs, dit fonds Barnier, Barnier, fortement mobilisé pour des opérations de construction résilientes, ainsi que la mobilisation financière de toutes les collectivités territoriales.

pour ce travail en bonne intelligence, dans la suite du rapport commun à leurs commissions, élaboré par nos collègues Jean François Rapin et Jean Yves Roux, sur les inondations ayant frappé l’ensemble du territoire durant l’hiver 2023 2024.

dans les cas d’aléas répétés ou de forte exposition aux aléas. Je salue également l’implication de notre collègue Pascal Martin, rapporteur pour avis,

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, en janvier 2020, je présentais ici même une proposition de loi visant à réformer le régime des catastrophes naturelles, que le Sénat votait à l’unanimité. Malgré la clairvoyance de notre Haute Assemblée, les députés lui ont préféré la loi Baudu, laquelle, bien que moins disante, tentait d’améliorer quelques points sur la question des franchises. Néanmoins, nous avons rapidement constaté ses insuffisances.

Outre ce temps précieux perdu, alors que la fréquence des catastrophes naturelles s’intensifie, il subsiste de nombreuses zones d’ombre pour garantir aux sinistrés une juste compensation et diffuser une culture du risque à tous les niveaux : préfectures, collectivités locales et particuliers.

Concernant le retrait gonflement des argiles, nous accueillons avec satisfaction les orientations du nouveau plan national d’adaptation au changement climatique présenté la semaine dernière,

La proposition de loi que nous examinons aujourd’hui apporte des évolutions bienvenues pour garantir l’intégrité du régime CatNat, qui repose sur des financements publics et privés.

ajouter une réassurance publique mutualisant les portefeuilles d’assurance au niveau national et bénéficiant de la garantie de l’État. Or la hausse très significative des catastrophes naturelles ne permet plus de répondre de manière satisfaisante aux demandes d’indemnisation.

Les articles 6 à 9 favorisent les assurés adoptant des mesures de prévention, qui pourront bénéficier de prêts à taux zéro, ainsi que les propriétaires de logements exposés aux risques naturels majeurs grâce au

En outre, une information régulière sur les catastrophes naturelles dans ces mêmes zones serait de nature à limiter les conséquences des sinistres, en ce qui concerne tant les dommages matériels que les accidents de personnes.

ces dossiers sont transmis par les préfets de département au ministère de l’intérieur. Ils sont alors présentés pour avis à une commission composée de représentants des différents ministères et d’experts techniques.

Les décisions portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, énumérant les communes reconnues et non reconnues, sont prises conjointement par le ministre chargé de l’économie et des finances, le ministre du budget et des comptes publics, le ministre de l’intérieur et, le cas échéant, celui de l’outre mer. Ces arrêtés interministériels sont publiés au. Il ressort donc de la loi et des différentes circulaires d’application que la procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle est largement déconcentrée et que la phase d’instruction des demandes à l’échelon ministériel vise seulement à garantir un traitement identique des situations communales sur l’ensemble du territoire national. Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est défavorable

Face aux nombreuses résiliations de contrats, après chaque sinistre climatique, particuliers, petites entreprises et collectivités sont déjà les premières victimes des catastrophes naturelles. Et pendant que les assurés peinent à se relever, les assureurs, eux, continuent de dégager des bénéfices, ce qui est complètement occulté dans notre discussion. En 2023,

Ce partage sera évolutif : en cas de hausse des coûts d’indemnisation liée à des événements climatiques plus fréquents, la répartition pourrait être revue pour s’adapter aux réalités économiques du secteur des assurances et à la charge assumée par les assurés.

pourront être appréciés. Afin de consolider les résultats définitifs de trois exercices, puis de réaliser les calculs et, enfin, de mettre en cohérence les résultats de ces calculs, une revalorisation du coefficient tous les cinq ans serait préférable.

telle mesure est nécessaire pour permettre aux assureurs de préparer leurs systèmes d’information et d’émettre les appels à cotisation annuels sans retard. Une annonce anticipée permet également aux assureurs de s’organiser efficacement et de garantir que les cotisations sont correctes dès le début de l’année suivante. Enfin, informer les assurés à l’avance renforce la confiance et la compréhension des changements tarifaires, assurant ainsi une gestion transparente et efficace des cotisations

2030 serait trop tardive au regard du besoin actuel de rééquilibrage financier du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles. De plus, les données relatives au coût de la sinistralité sur les dernières années existent déjà et montrent que le taux de surprime est actuellement trop

ce qui est souvent le cas, toutes les données intéressant le retrait gonflement des sols argileux, le fameux RGA, sont absentes du rapport d’expertise. Dans un tel cas, la cause du RGA n’étant pas identifiée, le rejet du dossier est certain.

Par ailleurs, le déclenchement du sinistre n’est pas exclusivement lié à la nature du sol. Il peut par exemple être causé par la présence de végétation aux abords immédiats de la construction ou la fuite de réseaux d’eau, qui qui induisent des mouvements rapides de retrait gonflement des couches argileuses. La réalisation systématique d’une étude géotechnique n’apporterait ainsi pas beaucoup d’éléments supplémentaires utiles

du bureau central de tarification (BCT). Au delà de la question de l’indemnisation, les personnes sinistrées expriment souvent la crainte de ne plus parvenir, à terme, à s’assurer de nouveau.

dans de nombreux cas, la renégociation des contrats d’assurance existants est aussi cruciale que la conclusion de nouveaux contrats. Elle permet d’ajuster la couverture assurantielle au plus près des besoins des assurés. L’impossibilité, dans la pratique, de renégocier

d’assurance couvrant les dommages aux biens, mais que ce n’est obligatoire que pour les locataires et propriétaires d’immeubles en copropriété. L’assureur peut refuser de conclure un tel contrat pour un motif autre

pour motif d’exposition au risque de catastrophe naturelle. En l’état actuel du droit, il appartient à l’assuré de prouver que le refus d’assurance est dû à la garantie catastrophe naturelle, ce qui est souvent difficile. Désormais,

fiable et opposable, laquelle n’existe pas à ce jour. Le dispositif implique également un encadrement strict des conditions d’activation de la présomption de refus, dans un contexte où le refus d’assurance peut résulter de nombreuses causes

Or notre modèle assurantiel est fondé sur la solidarité entre l’assuré et l’assureur. De plus, la mise en place d’une présomption de refus d’assurance ne préviendra pas les déserts assurantiels, qui empêchent de nombreux individus d’avoir accès à une assurance à

ce phénomène d’esquive, qui sera toxique à long terme pour l’universalité du régime assurantiel, doit être notre priorité. La stratégie qui consiste, pour certains assureurs, à fuir les zones les plus exposées, génératrices de pertes, pour mieux exploiter les zones à faible risque,

madame la ministre,

produisant une analyse impartiale des situations. Je vous rappelle en effet que cette commission émet un avis simple, qui ne lie pas l’autorité administrative, sur les 6 000 à 8 000 demandes communales déposées en moyenne chaque année. Elle se réunit pour cela entre quinze et vingt fois par an. Plusieurs mesures organisationnelles ont été prises ces dernières années, afin d’améliorer l’efficacité du dispositif. Ainsi, la dématérialisation de la procédure permet désormais à toutes les communes de France de déposer leurs demandes par internet en quelques minutes.

Ces progrès ne doivent pas être remis en cause par des contraintes organisationnelles nouvelles. Pour ce qui est de la transparence des décisions adoptées par la commission, je précise que celles ci sont fondées sur des critères et des méthodes d’analyse fixés par une circulaire du 29 avril 2024 pour l’ensemble des phénomènes naturels couverts par la garantie catastrophe naturelle. Cette instruction est opposable à l’administration et librement consultable sur le site Légifrance où est recensé Le point de vue des élus locaux sur l’ensemble du processus d’indemnisation et leur participation à la gouvernance générale du régime des catastrophes naturelles est en revanche indispensable.

pour déterminer la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, sur les conditions effectives de l’indemnisation des sinistrés, le délai, les montants d’indemnisation, les décisions de refus de prise en charge, ainsi que sur les modalités et les conditions d’intervention des experts d’assurance.

article 3, la loi Baudu était revenue sur les modulations de franchise qui frappaient les particuliers et les professionnels. C’était un bon début, qui avait d’ailleurs recueilli notre assentiment. Les collectivités territoriales et leurs groupements demeurent, quant à elles, soumises à des modulations significatives de leurs franchises lorsqu’elles n’ont pas adopté de plan de prévention des risques naturels.

L’instruction des dossiers suscite souvent un sentiment d’insatisfaction et d’incompréhension chez les sinistrés, notamment du fait de la part significative – plus de 50 % – des dossiers classés sans suite sur le territoire de communes pourtant reconnues en état de catastrophe naturelle.

Un décret visant à encadrer l’activité de ces experts spécifiquement pour le retrait gonflement des argiles doit être publié. Il doit, en particulier, donner une définition du contenu obligatoire attendu pour chaque rapport d’expertise.

et l’indépendance des expertises en matière de catastrophe naturelle, en apportant des garanties essentielles pour protéger le droit des assurés. Nous tenons compte également des dispositions de l’article 4, en soulignant la nécessité de reconnaître des qualifications particulières aux experts mandatés par les sociétés d’assurance. En effet, malgré les compétences nécessaires à l’exercice du métier d’expert, il n’existe actuellement aucune qualification minimale spécifique

pour garantir que les expertises soient menées par des professionnels qualifiés, indépendants et rémunérés de manière transparente, en nous appuyant sur des catégories existantes comme le tableau national des experts près le d’État. Les contrats qui lient les experts aux compagnies d’assurances posent parfois un problème d’indépendance. Une expertise neutre est essentielle pour garantir une certaine équité des décisions prises en cas de catastrophe naturelle ; cela ne passe pas uniquement par le lien contractuel. Nous souhaitons encadrer la sélection des experts en imposant des critères de compétence et d’indépendance, et en révisant leur mode de rémunération, afin de limiter les influences potentielles. l’avis de la commission

d’assurances. Même si le contrat qui lie l’expert à la compagnie d’assurances qui le mandate ne doit pas comporter de clauses d’intéressement, le contrat, par nature, crée un lien d’intérêt entre un client et un et un prestataire et n’assure pas la totale indépendance de l’expert. Pour rompre définitivement ce lien d’intérêt, il est souhaitable que les experts soient rémunérés par un fonds mutualisé et indépendant constitué par les compagnies d’assurances et géré paritairement entre représentants des compagnies d’assurances et représentants des assurés. Ce fonds n’est pas une dépense supplémentaire, puisqu’il est le fruit de la mutualisation des dépenses actuelles des compagnies d’assurances pour la rémunération des experts.

ne permettrait pas forcément de répondre à la problématique de l’indépendance des experts d’assurance. Les modalités de création de ce fonds nous paraissent imprécises à ce stade. Par ailleurs, le Gouvernement a déjà engagé des travaux portant sur l’encadrement de l’expertise d’assurance lors de sinistres, notamment en cas de retrait gonflement des argiles,

concrètement. L’assuré n’est souvent pas en mesure de disposer des informations nécessaires permettant d’établir les manquements aux nouvelles dispositions, les relations contractuelles entre personnes privées n’étant pas à la disposition du public. De plus, partie faible au contrat, l’assuré devrait porter un tel cas devant un juge civil pour être indemnisé du préjudice économique subi. Cela fait peser une charge probatoire trop importante sur les assurés. Ajouter une sanction pénale en cas de méconnaissance de ces nouvelles obligations obligations aurait un effet dissuasif certain et ouvrirait la porte à des poursuites qui ne pèsent pas uniquement sur les assurés. Par Par une simple plainte déposée ou sur le fondement du contrôle courant exercé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), les nouveaux principes seraient ainsi véritablement effectifs.

Monsieur Gontard,

Quel est l’avis du Gouvernement ? Le Gouvernement finalise actuellement les textes d’application de l’ordonnance du 8 février 2023 relative à la prise en charge des conséquences des désordres causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Cette ordonnance prévoit notamment un décret encadrant davantage les activités des experts en assurance chargés de procéder à l’établissement des expertises à la suite des sinistres ayant pour cause déterminante le retrait gonflement des argiles. Dans ce décret, qui devrait être publié d’ici à la fin de l’année – c’est quasiment brûlant, monsieur le

Cela étant dit, le principe d’une obligation d’affectation de l’indemnité d’assurance allouée après un sinistre lié à un RGA se justifie au regard des spécificités de ce péril, qui s’inscrit dans le temps long. Ce principe vise à responsabiliser les assurés et à éviter des sinistres de seconde génération. Le retour en arrière qu’entraînerait l’adoption de cet amendement nous paraît préjudiciable pour le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles. L’avis du Gouvernement est donc défavorable.

les sinistrés. Sur la question de la transparence de l’expertise, il est possible d’aller plus loin. Cet amendement vise donc à rendre automatique la communication des différents éléments de l’expertise aux deux parties du contrat.

initiale est transparente, moins elle est susceptible d’être contestée à l’occasion d’une contre expertise : le gain de temps et d’argent n’est pas négligeable. Mme Nadia Sollogoub. L’article A. 241 1 du code des assurances prévoyait que « l’assureur, sur le vu du rapport d’expertise préalablement communiqué à l’assuré, notifie à celui ci ses propositions définitives ». Cependant, les associations qui viennent en aide aux sinistrés victimes des phénomènes de retrait gonflement des argiles constatent que ces dispositions sont bien souvent contournées. Les assurés reçoivent davantage un rapport de constat du sinistre

Nous proposons ce faisant d’améliorer le processus de reconnaissance des catastrophes naturelles liées aux épisodes de sécheresse en y introduisant des critères supplémentaires, afin de rendre le dispositif plus fiable et plus complet. Actuellement, la reconnaissance d’un état de catastrophe naturelle de sécheresse repose principalement sur des critères météorologiques, comme le niveau d’humidité des sols superficiels. Ces critères sont certes pertinents, mais insuffisants,

pouvoir disposer d’un réseau météo agricole collectant en temps réel ces données, ce qui permettrait une analyse plus fine.

d’ordre juridique. De mon point de vue, l’amendement est aujourd’hui satisfait par une circulaire du ministère de l’intérieur du 29 avril 2024, publiée le 15 mai

les critères utilisés pour caractériser l’intensité anormale des épisodes de sécheresse et de réhydratation des sols, ont été en effet définies par une circulaire du 10 mai 2019, puis révisées par une circulaire du 29 avril 2024 pour prendre en compte les dispositions de l’ordonnance du 8 février 2023 relative à la prise en charge des conséquences des désordres causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.

et notamment les nouveaux critères utilisés pour caractériser l’intensité anormale des épisodes de sécheresse et de réhydratation des sols pour ce qui est des événements survenus à partir du 1 janvier 2024. La définition de la méthodologie par un décret n’est donc pas nécessaire. Par ailleurs, deux critères sont mis en œuvre de manière cumulative pour analyser la situation des communes un critère géotechnique fondé sur la présence d’argiles sensibles au phénomène de RGA sur le territoire communal ; d’autre part, un critère météorologique fondé sur l’analyse du niveau d’humidité des sols superficiels. Actuellement, pour établir ce niveau d’humidité des sols superficiels, les services de l’État s’appuient sur l’indicateur SWI (). Il s’agit d’un indice d’humidité des sols documenté dans la littérature scientifique et utilisé à l’échelle internationale. d’évaluer, sur une profondeur d’environ deux mètres, l’état de la réserve en eau du sol par rapport à la réserve utile : il s’agit en fait de l’eau disponible pour l’alimentation des plantes. Il prend en compte également de multiples facteurs : le niveau des nappes souterraines et des cours d’eau,

les résidences secondaires et les biens locatifs localisés en zone d’exposition forte et très forte, en instaurant pour ces seuls cas la liberté de fixation des primes et franchises d’assurance du régime d’indemnisation des catastrophes Cette proposition s’inscrit dans le droit fil du rapport Langreney, qui recommande de renforcer l’incitation à la prévention des risques pour ces catégories spécifiques.

En mars 2024, la question demeurait ouverte et la prise en charge des assureurs restait un sujet de préoccupation majeure. À l’heure actuelle, des délais différents coexistent dans le droit.

D’autre part, l’assurance doit verser l’indemnisation dans les trois mois qui suivent la date de remise effective de l’état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies.

du territoire. Cet amendement s’inscrit dans cette logique, notamment en reprenant une recommandation du rapport Langreney de 2023 qui prévoyait de « développer un mécanisme de nivellement des marges techniques entre zones à faible et forte exposition la modulation du prélèvement additionnel sur le régime CatNat au titre de la prévention Par ce rééquilibrage entre des zones à faible ou forte exposition, le but est à la fois d’empêcher la fuite des assureurs dans les cas de surexposition et de prévoir un nivellement tarifaire.

en droit aucun principe général d’obligation de reconstruction à l’identique. Au contraire, le principe est celui de la libre utilisation, par l’assuré, de la somme versée par l’assureur. En revanche, la combinaison de plusieurs dispositions du code des assurances conduit, en pratique, à privilégier les reconstructions à l’identique. Sans doute l’obligation

Cette solution à bénéfices multiples serait également favorable aux assureurs. Ceux ci, en effet, y gagneraient : l’augmentation de la valeur du bien après une reconstruction résiliente leur profiterait, dans le cas où le propriétaire chercherait à changer de contrat.

collègue, tend à intégrer dans le rapport d’expertise un rappel de l’absence d’obligation de reconstruction à l’identique.

en application de la loi Climat et Résilience, au mois d’avril 2023. Pour produire ces audits, il faut disposer d’une certification professionnelle de diagnostiqueur immobilier étendue à l’audit énergétique,

commune […] si cet épisode de sécheresse annuel intervient sur le territoire d’une commune limitrophe d’une commune ayant subi un épisode de sécheresse annuel anormal ou

Il est parfois difficile, pour un assuré qui n’est pas expert des catastrophes ni du code des assurances, de contester les conclusions d’un expert qu’il n’a pas choisi. Bien entendu, l’assuré peut demander une contre expertise, mais il devra la payer lui même et, de fait, les familles ou les petites entreprises touchées ont souvent du mal à mettre en œuvre cette faculté, notamment pour des raisons financières.

monsieur le rapporteur,

Mme la ministre déléguée. L’objet de cet amendement est de préciser le champ d’application de l’éco prêt à taux zéro (éco PTZ) destiné à financer des travaux de prévention du risque de retrait gonflement des argiles. Le Gouvernement a la volonté de faciliter le financement des travaux de prévention pour rendre le bâti plus résilient.

date d’entrée en vigueur de l’obligation de réalisation d’une étude sur le risque de retrait gonflement des argiles lors d’une construction. Nous souhaitons également préciser le champ des travaux de prévention finançables, établi sur la base des conclusions

Actuellement, la rénovation énergétique de logements fortement exposés aux risques naturels et pour lesquels n’est prise aucune mesure de prévention représente

J’entends, au regard des principes constitutionnels permettant d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics, que l’on souhaite conditionner les aides à la rénovation énergétique à la réalisation de travaux de prévention des risques, mais il serait souhaitable de faire preuve, en la matière, d’un peu de logique. De fait, par ce conditionnement, les ménages les plus précaires dont le logement serait exposé aux risques naturels majeurs verraient s’ajouter à ce risque une précarité énergétique accrue. En effet, comment les ménages n’ayant pas la capacité financière de mettre en œuvre des travaux de rénovation énergétique auraient ils davantage les moyens financiers d’exécuter des travaux de dérisquage ? Ce conditionnement risquerait de retirer des millions de biens du marché de la rénovation énergétique et, ainsi, de créer un manque à gagner important pour les acteurs du secteur, en plus d’aggraver notre retard en matière de transition écologique. Enfin, cette obligation enjointe aux particuliers ne bénéficie pas de la même valeur lorsqu’il s’agit de la commande publique : les élus locaux sont régulièrement sommés d’utiliser leurs primes d’assurance pour effectuer des reconstructions à l’identique, alors même que le bien endommagé aurait pu être amélioré, notamment sur le plan de la prévention des risques naturels. Pourtant, il n’existe pas en droit de principe général d’obligation de reconstruction à l’identique… Pour Pour ces raisons, nous estimons que conditionner les aides à la rénovation énergétique à la réalisation de travaux de prévention des risques n’est pas la solution. Au contraire, ce serait un facteur d’immobilisme tant pour notre adaptation au dérèglement climatique que pour notre transition écologique.

Toutefois, la mise en place d’un conditionnement de l’aide MaPrimeRénov’ à la réalisation de travaux de prévention lorsque le logement se situe dans une zone d’exposition élevée à un ou plusieurs risques naturels majeurs ne saurait intervenir à court terme sans une formation et une préparation suffisantes de l’ensemble des acteurs de l’écosystème de la rénovation énergétique. À défaut, les auteurs de ces deux amendements, cette exigence ne ferait que diminuer le nombre de rénovations énergétiques sans pour autant accroître significativement le nombre de travaux de prévention. En conséquence, le Gouvernement propose, dans un premier temps, de privilégier l’information et la sensibilisation des en intégrant à leur accompagnement dans un parcours de rénovation globale le repérage des risques constructifs associés au phénomène des mouvements de terrain liés au retrait gonflement des argiles.

ne devrait pas intervenir à court terme sans une préparation suffisante de l’ensemble des acteurs. De fait, 10 millions de maisons individuelles pourraient être concernées par un tel conditionnement, qui risquerait d’avoir pour effet de réduire le rythme de rénovation énergétique sans accroître la prévention. Des travaux d’expertise doivent être menés pour mieux évaluer l’effet de cet éventuel conditionnement. Le Gouvernement propose, dans un premier temps, de privilégier l’information et la sensibilisation des ménages, en renforçant dès à présent le corpus de formation des conseillers pour y ajouter une mission d’accompagnement au repérage des risques constructifs.

à ce que l’accès à MaPrimeRénov’ reste ouvert aux propriétaires, notamment les plus modestes, qui ont un besoin urgent d’engager des travaux de rénovation énergétique. L’article 8 risque de rendre l’accès à cette aide plus difficile pour beaucoup de foyers,

la réalité structurelle de chaque logement, et non seulement la zone géographique où il se trouve. Ce ciblage éviterait que les propriétaires soient privés de MaPrimeRénov’ au seul motif que leur logement se situe dans une zone classée à risques, alors même que son état ne le rend pas directement vulnérable à une catastrophe.

Cet amendement tend à décaler d’une année l’entrée en vigueur du conditionnement de MaPrimeRénov’, pour les logements les plus exposés aux risques naturels majeurs, à la réalisation de travaux de prévention des risques. Ce report d’un an permettrait de subordonner son application aux conclusions du rapport que le Gouvernement devra remettre au Parlement dans le délai d’un an suivant la promulgation de la présente loi, évaluant l’incidence du conditionnement de la prime de transition écologique à la réalisation de travaux de prévention des risques pour les logements les plus fortement exposés exposés aux risques naturels majeurs. En effet, une telle mesure pourrait avoir des incidences non négligeables, tant économiquement, par le manque à gagner qu’elle engendrerait pour les acteurs de la rénovation énergétique, qu’environnementalement, du fait du retard

Le présent amendement fait écho à celui que j’ai présenté à l’article 8. Il vise à compléter la mission d’accompagnement à la rénovation énergétique assurée par les structures agréées « Mon Accompagnateur Rénov’ en y incluant une assistance au repérage des risques constructifs associés au phénomène de retrait gonflement des argiles. Cette nouvelle mission sera réalisée au bénéfice des logements situés dans une zone d’exposition moyenne ou forte à l’aléa de retrait gonflement des argiles. Elle permettra d’accompagner les ménages souhaitant s’engager dans un projet de rénovation d’ampleur dans le repérage des risques de sinistres liés au retrait gonflement des argiles et la mise en

de mieux prévenir les catastrophes naturelles futures et de limiter leurs impacts, qu’ils soient financiers, infrastructurels ou humains. Ainsi convient il de profiter des travaux de réparation à conduire sur le parc immobilier des collectivités sinistrées par des catastrophes naturelles pour réfléchir à leur adaptation face à ces risques. On le sait, les instructions d’urbanisme et les autorisations environnementales

En d’autres termes, en voulant élargir un dispositif qui fonctionne bien, on va menacer son efficacité. On sait que le phénomène de RGA touche à lui seul près de 50 % du territoire métropolitain et affecte spécifiquement les particuliers, là

Le fonds Barnier a vocation à financer la prévention des risques naturels majeurs, c’est à dire des phénomènes brutaux présentant une menace grave pour les vies humaines, alors que le RGA est un phénomène lent et progressif, dont les conséquences se manifestent après une série de cycles naturels. Le RGA est avant tout dû à un défaut de conception du bâtiment. Le Gouvernement travaille donc à identifier les solutions les plus efficaces et les plus durables pour résoudre ce problème majeur pour les bâtiments existants.

Madame Lavarde,

Le présent amendement vise à donner aux collectivités locales la possibilité d’intégrer le risque de RGA dans les documents d’urbanisme qu’elles élaborent. Les orientations d’aménagement et de programmation s’imposant à la délivrance de toute autorisation d’urbanisme, la collectivité pourrait ainsi agir sur la résilience du bâti existant en renseignant les propriétaires de parcelles sur les travaux de prévention à réaliser. Concernant les nouvelles constructions, ce nouvel outil permettrait d’améliorer les conditions d’implantation et les méthodes de construction en demandant, selon la gravité du risque détecté, des obligations spécifiques telles que la réalisation d’un diagnostic G2 Pro ou encore d’un diagnostic horizontal. Une telle mesure participerait à la diffusion à l’échelle locale d’une nécessaire culture du risque, à l’heure où des solutions techniques émergent et confirment leur pertinence face au RGA.

Madame la sénatrice, votre amendement tend à intégrer la prise en compte du risque de retrait gonflement des argiles dans les orientations d’aménagement et de programmation des plans locaux d’urbanisme. Or ce risque est déjà bien pris en compte dans les dispositions du code de l’urbanisme et dans les documents de planification. En effet, En effet, la prévention des risques naturels prévisibles fait partie des objectifs généraux de l’urbanisme que l’action des collectivités publiques doit viser. Par ailleurs, si le risque de retrait gonflement des argiles est identifié au sein d’un plan de prévention des risques naturels, il aura valeur d’une servitude d’utilité publique qui devra être annexée au plan local d’urbanisme. Dans ce cas, les prescriptions liées à ce risque s’imposeront aux règles du plan local d’urbanisme. Les orientations d’aménagement et de programmation seront également définies en tenant compte des risques identifiés sur le territoire de la commune. Si ce risque n’est pas encore défini en tant que servitude d’utilité publique, la collectivité peut déjà le prendre en compte dans le plan local d’urbanisme et délimiter des secteurs où l’implantation de constructions est soumise à conditions ou interdite. Il n’est donc pas utile de le repréciser parmi les possibilités offertes aux orientations d’aménagement et de programmation. Pour ces raisons, cet amendement étant satisfait, j’en demande le retrait.

Cependant, le fait qu’un phénomène soit inédit et peu étudié ne saurait constituer un argument valide pour ne pas le considérer comme une catastrophe naturelle,

Faute de financement approprié et dédié de manière pérenne, c’est la DETR qui finance le ramassage et le traitement des sargasses, ce qui n’est pas normal. Quel est l’avis de la commission

cet amendement ne nous semble pas constituer une réponse appropriée,… Ah ! … car il remet en cause le fondement du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles. La définition d’une catastrophe naturelle a été strictement encadrée dès la création du régime et repose en premier lieu sur la reconnaissance du caractère d’intensité anormale du phénomène. Revenir sur cette définition reviendrait à déstabiliser l’ensemble d’un système qui a prouvé maintes fois sa pertinence. Pour ce qui est des sargasses, ce n’est pas le caractère nouveau de l’échouage massif

de causalité entre le phénomène et les dégâts recensés qui explique d’abord le rejet des demandes communales de reconnaissance. Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable

Les ouvrages d’art n’étant pas assurés, ils n’ont pas à entrer dans le périmètre du fonds Barnier. Le financement des réparations et des reconstructions des ouvrages d’art après une catastrophe naturelle relève de la dotation de solidarité aux collectivités victimes d’événements climatiques ou géologiques, la DSEC, pour ce qui est des ouvrages relevant des collectivités territoriales.

nous –, permettrait de renforcer les actions de prévention tout en protégeant la biodiversité, enjeu crucial face au défi climatique. Les solutions fondées sur la nature, telles que la reforestation ou la création de barrières naturelles, sont évidemment à privilégier, compte tenu de leur durabilité et de leur impact positif en matière de biodiversité et de gestion de l’eau notamment. Elles réduisent les impacts des catastrophes naturelles, améliorent la résilience des territoires et contribuent à la conservation de la biodiversité.

l’avis du Gouvernement ?

Monsieur le sénateur, vous proposez d’assouplir les conditions de mobilisation du fonds Barnier pour les territoires ultramarins sans remettre en cause les règles en vigueur pour l’Hexagone. Les territoires ultramarins qui relèvent du code de l’environnement sont éligibles au fonds Barnier comme le reste du territoire national. Je vais vous citer deux exemples significatifs de l’engagement de l’État et de la forte mobilisation du fonds Barnier outre mer. En premier lieu, pour tenir compte de l’extrême exposition des Antilles au risque sismique, des dispositions spécifiques du fonds existent pour réduire le risque d’effondrement de certains bâtiments, comme les écoles ou les bâtiments des services d’incendie et de secours, dans le cadre du plan Séisme Antilles. En second lieu, le village de Miquelon, très exposé aux risques de submersion marine, va entamer à partir de 2025 une délocalisation qui sera financée également à l’aide du fonds Barnier. En moyenne, la mobilisation est de 3 euros par habitant sur le territoire national contre 22 euros en outre mer. Cette forte outre mer. Cette forte utilisation, légitime du fait de la forte exposition des territoires ultramarins aux risques naturels majeurs, démontre la bonne utilisation du fonds Barnier et son adéquation de ces territoires. Le fonds Barnier reposant sur le principe de solidarité nationale, il ne me semble pas souhaitable de différencier, au delà de ce qui existe déjà pour le cas spécifique du risque sismique, ni les règles de mobilisation du fonds ni les taux de subvention applicables. C’est pourquoi j’émets un avis défavorable

la dotation de solidarité en faveur des équipements des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques, il y a quelques années,

opérationnelles importantes. À l’occasion de la vente d’un terrain constructible, les détails de conception d’une future construction ne sont que très rarement connus. Il n’est donc guère possible de réaliser à cette étape une étude géotechnique de conception, par rapport à l’étude géotechnique préalable exigée dans le droit en vigueur. De même, les plans de la construction sont susceptibles d’être ajustés postérieurement à la signature du contrat de construction d’une maison individuelle, nous le savons tous. Il apparaît donc nécessaire de laisser de la souplesse à cette étape, d’autant plus qu’une étude G2 est bien plus coûteuse coûteuse et contraignante. Avant tout renforcement des exigences, il est nécessaire de disposer d’un retour d’expérience sur l’efficacité de la mise en œuvre des mesures de la loi Élan visant à garantir la résilience des constructions neuves face au risque de RGA. l’avis de la commission

repose essentiellement sur les assurés, sans impliquer suffisamment l’État, au travers du fonds Barnier, et les assureurs. Toutes les études aboutissent à la conclusion que les pouvoirs publics n’anticipent pas assez les politiques et les investissements nécessaires à l’adaptation et qu’ils ne protègent pas à ce jour, les citoyens contre le réchauffement climatique, faute de politique globale ambitieuse à la hauteur du défi à relever. Selon les scientifiques, réduire les gaz à effet de serre ne coûterait que le quart du coût des dommages que le changement climatique pourrait nous infliger, soit un retour sur investissement d’au moins 4 pour 1. Malheureusement, alors que nous devrions accélérer nos efforts en matière de transition écologique, nous déplorons que le Gouvernement ait fait le choix de restrictions budgétaires,

l’équilibre du système uniquement sur l’effort des assurés, nonobstant les autres responsabilités dues à l’accélération des dérèglements climatiques. Pour conclure, je citerai au besoin de production, il convient d’opposer un impératif de défense de l’habitabilité de la planète. Pour nous, écologistes, c’est la priorité numéro un des politiques publiques. S’il faut traiter la remédiation et l’adaptation au réchauffement climatique un modèle de financement mieux adapté et plus juste, il importe, plus que jamais, d’investir dans des politiques d’atténuation ambitieuses, avec comme ligne de mire la neutralité carbone en 2050. C’est ainsi,

très largement en faveur de cette proposition de loi. Très bien ! Je profite de cette occasion pour saluer et féliciter toutes celles et tous ceux qui s’impliquent et s’engagent en faveur d’une meilleure prise en charge de nos concitoyennes et de nos concitoyens qui traversent ces catastrophes de nature à bouleverser leur vie.

Le scrutin est clos.

La séance est levée.